monsieur le président.

La situation actuelle liée à l'épidémie du Covid-19 impose de prendre des décisions de bon sens économique. Notre pays doit conserver, si ce n'est récupérer, une souveraineté sanitaire. Notre dépendance vis-à-vis de l'Asie est devenue insupportable et préjudiciable, la crise sanitaire actuelle l'atteste. En effet, après la pénurie de masques, de tests de dépistage et de médicaments il y a quelques semaines, nous ne pouvons que constater que la France est totalement dépendante et extrêmement fragilisée sur le plan sanitaire, ce qui représente un véritable danger pour la santé de nos concitoyens. L'entreprise Luxfer est la seule en Europe à fabriquer des bouteilles d'oxygène. Aujourd'hui, nous ne connaissons pas l'état des stocks en France. Or ces bouteilles seront certainement utiles dans les jours et mois qui viennent. La société Famar est spécialisée dans la production pharmaceutique, en particulier de la nivaquine, un antipaludique à base de chloroquine, qui est l'une des molécules dont l'utilisation est envisagée sérieusement pour le traitement du Covid-19, notamment en phase initiale de la maladie. La société, installée près de Lyon, est actuellement en redressement judiciaire. Il est essentiel de veiller, eu égard aux enjeux, à ce qu'elle ne soit pas liquidée ou reprise par un fonds vautour qui spéculerait sur le prix de vente de cette molécule ou par un repreneur qui chercherait à en délocaliser la production. Il est urgent de procéder à la réquisition et à la nationalisation des entreprises Luxfer et Famar, afin d'assurer la souveraineté française et européenne en matière de fabrication de bouteilles d'oxygène. Il est nécessaire de préparer leur réouverture avec des capitaux publics. La parole est à M. Pascal Savoldelli,

après l'amendement adopté par le Sénat -, qui permet de prendre des participations dans des entreprises. Il s'agit du programme « Plan d'urgence face à la crise sanitaire et renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

de soutenir mon collègue Jean-Yves Leconte sur la couverture santé. Peut-être divergerons-nous sur les montants nécessaires, mais la réalité est que nous aurons besoin d'une aide exceptionnelle, qu'il est important d'ouvrir au plus vite. À l'étranger, les conseils consulaires pour l'aide sociale (CCPAS) se réunissent une fois par an,

En effet, la majorité de ces Français ne sont pas des expatriés détachés par l'entreprise pour un contrat limité : ils sont salariés dans des entreprises locales, autoentrepreneurs, professeurs vacataires dans les instituts français et les alliances françaises ou travaillent dans le tourisme et le commerce en contrats

Cette aide exceptionnelle pourrait les aider à suivre une formation, par exemple pour se reconvertir et trouver un emploi dans un secteur plus porteur, à payer une location pour ne pas se retrouver pas à la rue ou à payer des frais médicaux s'ils ont perdu leur couverture médicale en perdant leur emploi.

Ouvrons ces crédits, afin que les CCPAS soient en mesure de répondre aux demandes du 1,8 million de Français inscrits dans nos consulats. Quel

pour accompagner les entreprises, mais aussi pour vérifier que les dispositifs préconisés sont effectivement mis en oeuvre par les employeurs, afin de préserver la santé

dispose que seules les entreprises sont concernées par le dispositif de prêt garanti par l'État ; les sociétés civiles immobilières (SCI) en sont expressément exclues. Les monuments historiques recevant du public et détenus en nom propre ou en SCI sont pourtant fortement affectés par les mesures de confinement de confinement ; ils ne génèrent de revenus que grâce à l'accueil du public, sous toutes ses formes. Par ailleurs, les modalités d'application du dispositif du mécénat affecté aux monuments historiques privés imposent que les éventuels bénéfices soient affectés exclusivement aux travaux, ce qui

L'Institut de recherches économiques et sociales a mis en lumière le fait que certains enfants n'ont bien souvent pour tout repas équilibré dans la journée que celui qu'on leur sert à la cantine de l'école. De plus, selon l'Insee, sur les 8 millions d'enfants qui fréquentent les cantines scolaires, 14,2 % sont issus de familles vivant sous le seuil de pauvreté. Chaque enfant doit avoir le droit de s'alimenter convenablement, qui plus est dans le cadre scolaire, et ce sans que le budget de sa famille ne soit un obstacle. L'objet de cet amendement est donc d'ouvrir des crédits,

les hommes déclarait au : « Je crée un fonds spécial financé par l'État d'un million d'euros, pour aider les associations de terrain à s'adapter à la période.

Dans cette logique, nous proposons de transférer 1 million d'euros, sur les 7,5 milliards d'euros prévus pour le fonds de solidarité, à un nouveau fonds d'urgence de lutte contre les violences intrafamiliales. Quel

explique ce qu'elle fera de ce million d'euros : « Acheter du matériel de télétravail, soutenir les déplacements en taxi, préparer la reprise. Nous finançons jusqu'à 20 000 nuitées d'hôtel, pour que les femmes, pendant le confinement, puissent fuir un homme violent, et aussi pour écarter immédiatement du domicile des conjoints violents. » Je suis en train non pas de préparer l'avenir, l'avenir, mais de donner les moyens de répondre à l'augmentation spectaculaire des violences contre les femmes qui se produit actuellement : j'entends vous permettre

En l'occurrence, madame Rossignol, contrairement à vous peut-être, il m'est arrivé de diriger une collectivité locale et d'avoir à gérer quotidiennement les problèmes que vous évoquez.

pour le produit des amendes des radars, la philosophie du dispositif étant que les infractions financent la prévention. Les radars financent les radars : dans cette logique, nous fonctionnons en circuit fermé, avec un mécanisme qui fait que plus le produit des amendes est important, plus le compte d'affectation est doté d'un budget élevé, plus l'entretien et l'installation de nouveaux radars vont pouvoir se multiplier. Il y a un effet exponentiel. L'idée est d'aller vers une logique similaire dans la santé. Compte tenu des risques que font encourir au personnel soignant les gens qui ne respectent pas le confinement,

en commission des lois jeudi dernier ; il s'est déclaré ouvert à l'idée d'une affectation symbolique du produit des amendes. Nul doute que le Gouvernement dispose de tous les moyens techniques pour ce faire. Aussi, l'adoption de cet amendement d'appel ne saurait que l'encourager à avancer résolument dans cette voie. Je vais retirer cet amendement, monsieur le président, mais j'aimerais avoir le sentiment du ministre par rapport

cela nous semble insuffisant pour pallier, notamment, la perte d'un stage gratifié ou d'un emploi pour près de la moitié d'entre eux. Or, chacun le sait ici, les étudiants sont actuellement largement exclus des plans d'aide

et développées urgemment et massivement. Il s'agit d'apporter à la nation une autre issue que le confinement, qui risque d'être imposé périodiquement à la population française s'il n'est pas possible de trouver des moyens efficaces de lutter contre le virus. Aussi, afin de donner sans tarder les moyens budgétaires dont la communauté de la santé et de la recherche a besoin, cet amendement, contraint par les normes constitutionnelles imposées par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), a pour objet d'apporter sans attendre aux programmes 150 et 172 de la mission interministérielle « Recherche et enseignement supérieur

Mme Éliane Assassi. Pour la première fois en soixante-dix ans, Emmaüs a lancé un appel aux dons financiers pour collecter 5 millions d'euros et survivre. L'association, qui aide 20 000 personnes parmi les plus fragiles en France, fait face aujourd'hui à un arrêt total de son activité et donc à une disparition complète des dons en nature qui font son budget. Ne restent aujourd'hui que 79 des 289 structures en mesure d'aider les sans-abri, les chômeurs de longue durée, les familles surendettées, les réfugiés et les personnes sortant de prison en réinsertion ou encore les gens du voyage, qui ont besoin d'aide. Sans cet apport de dons, c'est un pilier de la solidarité nationale qui pourrait disparaître, d'autant plus que les grands événements de l'association, qui peuvent constituer 40 % des budgets fédéraux, sont d'ores et déjà annulés.

printaniers généralement sources de revenus. J'ai évoqué Emmaüs, mais j'aurais pu citer d'autres associations caritatives comme le Secours catholique ou le Secours populaire. Quant aux associations qui ont maintenu leur activité, elles se retrouvent aujourd'hui submergées par les demandes de leurs bénéficiaires.

Évidemment, nous soutenons la reconnaissance du travail des personnels de santé et des personnels administratifs, qui ont travaillé sans compter leurs heures en revalorisant leur salaire.

Pourtant, c'est bien l'ensemble des personnels qui s'est mobilisé, y compris dans des établissements dits « de deuxième ligne », pour accueillir les malades transférés des établissements de première ligne. Surtout, ces primes vont aggraver le déficit de la sécurité sociale, en raison des exonérations de cotisations sociales, comme nous avons eu l'occasion de vous le rappeler avec notre amendement de compensation intégrale des exonérations par l'État. Notre amendement vise donc à maintenir les primes

de court terme pour l'ensemble des personnels soignants comme pour l'ensemble des fonctionnaires mobilisés, afin de majorer les heures supplémentaires effectuées sous forme de prime exceptionnelle ». En temps d'urgence sanitaire, où le confinement a constitué notre principale arme contre le virus, les 122 000 infirmiers libéraux ont intensifié leurs déplacements à domicile aux fins de prendre soin des malades du Covid-19. Ce sont aussi les infirmiers libéraux qui ont permis le maintien d'un suivi médical minimal pour les personnes faibles, malades et isolées, qui n'ont plus accès aussi facilement à leur médecin. Pourtant, leur rémunération horaire est passée de 12,5 euros à seulement 15 euros, et cela uniquement pour les consultations de patients positifs au Covid-19 ou suspectés de l'être. Cet amendement vise donc à faire bénéficier les infirmiers libéraux de la prime exceptionnelle réservée aux aides-soignants de l'hôpital. Pour lutter contre ce virus, l'ensemble de nos forces médicales est mobilisé ; il doit donc être gratifié sans inégalités. Quel

Il est difficile de comparer avec les infirmiers libéraux, qui, eux, ont parfois exposé leur vie en étant au contact des patients. Je comprends que des mesures soient prises pour venir en aide aux professions libérales qui ont été totalement déstabilisées, mais le cas des infirmiers libéraux entre bien dans un champ différent.

à l'intérieur d'une entreprise, sans les interdire. Il existe actuellement des dispositifs de plafonnement dans les entreprises publiques. Nous proposons que, au-delà d'un écart de 1 à 20 entre le plus faible et le plus élevé des salaires, il n'y ait plus de déductibilité des charges de

du même niveau d'avantage fiscal qui est pratiqué dans les autres départements d'outre-mer pour les opérations de rénovation hôtelière. Compte tenu de la crise qui frappe le secteur du tourisme et de l'hôtellerie outre-mer, et alors que Saint-Martin est aujourd'hui encore un territoire en reconstruction, ayant besoin d'incitations financières pour attirer les investisseurs et procéder aux rénovations hôtelières il n'y a désormais aucune justification au fait que cette collectivité subisse un taux minoré par rapport à celui qui est applicable dans les autres départements d'outre-mer. Pour rappel, cet amendement avait été adopté au Sénat avec un avis de sagesse, dans le cadre du PLF pour 2020, avant d'être supprimé par l'Assemblée nationale.

Cet amendement tend à déplafonner les dons en nature. La crise actuelle a un impact très fort sur les ventes, notamment de fromages AOC Elle fait peser une lourde menace sur ces filières, qui voient leurs chiffres d'affaires diminuer et éprouvent des difficultés à écouler leurs stocks. En effet, les produits laitiers AOP et IGP sont commercialisés chez les

Cet amendement vise à corriger cette situation en déplafonnant les dons, en leur permettant de bénéficier d'une réduction d'impôt équivalant à 60 % du coût de revient du produit. Il a donc une forte dimension économique, mais également sociale.

Les entreprises qui pourraient bénéficier de cette exonération sont celles qui sont concernées par l'obligation de fermeture ou par une diminution d'au moins 25 % de leur chiffre d'affaires. Dans les territoires ruraux, une telle disposition serait un moyen pour les communes d'aider leurs commerçants, restaurateurs, hôteliers, petits entrepreneurs ou encore artisans, qui font vivre leur territoire et dont la pérennité est bien souvent menacée.

La délibération devant être de portée générale, toute entreprise entrant dans les critères d'éligibilité définis dans le cadre de la délibération pourrait ainsi bénéficier de cette exonération, ce qui écarterait le risque de rupture d'égalité. Quel

reprendre un dispositif mis en place par le gouvernement Jospin en 2000, sous le septennat de Jacques Chirac. Il n'y a donc là rien d'inédit. Concrètement, il s'agit de permettre aux entreprises des départements, territoires et régions d'outre-mer, de demander un moratoire pour le paiement de leurs dettes sociales pendant un an. Par ailleurs, un abandon partiel des dettes sociales pourrait être consenti aux entreprises, dans la limite de 50 %. Compte tenu des spécificités caractérisant souvent les économies ultramarines, faites d'entreprises subissant aléas climatiques- sargasses, cyclones, etc. -, et fortement sujettes aux crises conjoncturelles, l'adoption de cet amendement de bon sens permettrait de favoriser utilement la reprise d'activité en période post-crise.

permettre aux entreprises de bénéficier d'un plan d'apurement de leur dette fiscale. Cet amendement a donc pour objet la suspension de droit pour une période de six mois des poursuites et des mesures de recouvrement forcé des dettes fiscales antérieures au 1janvier 2020.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme les plus observateurs d'entre vous auront pu le noter,

le Président de la République a eu raison d'indiquer que l'ensemble des mesures de lutte contre la crise sanitaire à laquelle nous sommes confrontés doivent être prises « quoi qu'il en coûte quoi qu'il en coûte ». Cela signifie que tout cela n'est pas gratuit, que cela a un prix, et qu'il faut bien en assurer le financement. Il existe plusieurs façons de financer.

Il n'est pas interdit de se poser des questions sur la manière de financer les dépenses que l'on engage, ni peut-être de s'interroger sur la manière dont les choses ont été faites depuis 2008. À court terme, j'en conviens, monsieur le ministre, un certain nombre de chiffres allaient dans le bon sens.

une taxe sur le capital au niveau mondial, nous aurons un vrai problème concernant le maintien de l'autonomie stratégique de nos pays. En effet, financer la dette en faisant en sorte qu'elle ne coûte pas cher,

l'année suivante. Pour cette année, cela aurait dû se faire en octobre 2019. En raison de la situation économique liée à l'épidémie du Covid-19, certaines collectivités souhaiteraient faire profiter de cet abattement leurs commerces, en particulier de centre-ville. Il est donc proposé ici de rouvrir le délai permettant aux collectivités territoriales et aux EPCI de voter cet abattement. Je connais maintenant la dextérité de Bercy ! Il ne devrait donc pas y avoir de problème pour procéder à cet est à M. le rapporteur général.

sont concentrés sur les urgences actuelles. Je le souligne, l'efficacité de ces services a été démontrée ces derniers jours. En revanche, il est possible pour les collectivités locales de moduler le taux jusqu'au 3 juillet,

Dans le droit actuel, aucune disposition ne les autorise à donner mandat à un tiers d'exécuter leurs dépenses ou leurs recettes. Cela pose des difficultés dans plusieurs situations, notamment lorsque les fonds sont récoltés par le

est l'avis du Gouvernement ? Cela a été dit, il s'agit d'élargir ce qui existe déjà pour des établissements publics nationaux et des collectivités locales. Cela fonctionne bien, et c'est le bon moment pour les hôpitaux.

démarches consécutives à un décès. Au nombre de celles-ci figure l'enregistrement de la déclaration de succession, qui doit intervenir dans un délai de six mois. Or la réduction des activités postales, la fermeture de certaines études notariales, la limitation des déplacements et le fonctionnement au ralenti

cette même période, prévoit que les adaptations des délais « ne s'appliquent pas aux déclarations servant à l'imposition et à l'assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts, droits et taxes ». Afin de ne pas ajouter des pénalités financières à des situations humainement difficiles, il est proposé dans cet excellent amendement de suspendre ce délai de six mois pour l'enregistrement des déclarations de successions

à permettre aux contributeurs privés, avec des mesures fiscales incitatives pour 2020, de participer aux recettes du fonds de solidarité mis en place par l'État.

je veux rappeler que le niveau de l'aide fiscale pour les dons des particuliers en faveur des organismes d'aide aux personnes en détresse est déjà très favorable, puisque l'État prend en charge les trois quarts du montant du don, dans la limite de 552 euros par versement, et les deux tiers au-delà de ce plafond.

par les entreprises au profit des organismes éligibles, et pas uniquement de ceux que vous visez, a été doublé par la loi de finances : il est passé de 10 000 à 20 000 euros. Monsieur Retailleau,

Le cahier des charges qui a été adopté pour appliquer l'article 6 de la première loi de finances rectificative exclut les SCI qui gèrent des monuments historiques ouverts au public de l'accès aux prêts garantis par l'État. Ces monuments, comme les autres structures culturelles, sont pourtant les premières victimes économiques d'un confinement qui pourrait être appelé, les concernant, à durer au-delà du 11 mai. Dans mon département, je veux citer l'exemple du château de Vaux-le-Vicomte, qui emploie quatre-vingts salariés- c'est donc une vraie entreprise

sur ce type de site, fragilisant les recettes de billetterie. Il ressort des échanges entre le Gouvernement et le rapporteur général de la commission des finances que la nouvelle rédaction proposée pour le présent article 7 permettrait de lever toute ambiguïté et de faciliter le financement de ces structures. M. Le Maire a même jugé devant l'Assemblée nationale

J'espère, madame la secrétaire d'État, que vous pourrez confirmer cette ouverture et nous indiquer que le cahier des charges sera rapidement modifié. Ce cahier des charges ne devra pas viser que les seules SCI commerciales, il devra également permettre aux propriétaires en nom propre d'accéder à ce dispositif, car une grande majorité des monuments historiques ouverts à la visite ou accueillant du public sous différentes formes- chambres d'hôte, location pour des réceptions, etc. -sont en effet gérés de cette façon, sans structure civile.

amendement vise à autoriser les intermédiaires en financement participatif (IFP) à distribuer des prêts garantis par l'État. Cette distribution s'inscrira dans le cadre défini entre l'État, BPI et la place, dans le respect du cahier des charges et des procédures définies par arrêté du ministre chargé de l'économie et dans un cadre d'égalité concurrentielle avec les établissements de crédit et les sociétés de financement. les sociétés de financement. Les IFP étant tenus à des obligations de bonne conduite vis-à-vis des prêteurs en vertu du code monétaire et financier, l'amendement a pour objet que la responsabilité de l'IFP est engagée vis-à-vis des prêteurs, en cas de défaut de l'emprunteur et d'appel à la garantie de l'État et dans l'hypothèse où le prêt proposé l'intermédiaire ne répondrait pas aux critères d'éligibilité applicables. Ce risque a vocation à être couvert par le contrat d'assurance souscrit par l'IFP contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile Il sera également précisé au niveau réglementaire ou infraréglementaire que les IFP assureront la notification des prêts à BPI après avoir vérifié le respect du cahier des charges et que les prêts garantis par l'État seront tarifiés de manière responsable, à prix coutant pour la plateforme et à un taux modéré pour les prêteurs individuels.

Rappelons que ces entreprises, même si elles ne sont pas immatriculées en France, participent à notre rayonnement économique et culturel et bénéficient à ce titre des dispositifs de développement de la French Tech à l'étranger, notamment.

de monuments historiques classés ou inscrits et qui collectent des recettes liées à l'accueil du public, quel que soit le régime d'imposition de la SCI- le champ d'application est donc large. S'agissant des entrepreneurs individuels, ils sont d'ores et déjà couverts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

certes minoritaires, dans lesquels nous n'avons pas de solutions. C'est la raison d'être de l'amendement de la commission des finances, qui n'est sans doute pas parfait, mais qui offre une alternative au dispositif de prêts par les banques et par le fonds

de prendre les 10 % de risques qui ne sont pas couverts, la plupart des demandes de prêts se situant au-dessous de 150 000 euros et émanant de petites entreprises éligibles au taux maximal de garantie de 90 %. Il est donc proposé d'ouvrir une exception, même si le dispositif

En effet, la suppression de la mention de l'article qui exclut ces entreprises a été assortie de la modification de l'arrêté d'application du PGE, afin d'inclure uniquement les entreprises qui ont entamé une procédure collective en 2020. Nous pensons au contraire qu'il faut soutenir ces entreprises, qui ont entamé des procédures collectives depuis plusieurs mois et qui, après ces efforts, commencent à se rétablir.

accordés aux entreprises avec la garantie de l'État. En effet, il serait malvenu que ces établissements en viennent à appliquer des taux excessifs, alors que l'objet de ces prêts est de soutenir l'économie en période de crise. Cette contrainte d'encadrement doit être mise en parallèle avec la garantie accordée par l'État de 70 % à 90 %. Quel

15 avril 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020.

les contours de l'éligibilité à ce PGE mériteraient d'être encore précisés et renforcés. Pourquoi ne pas l'ouvrir à certaines entreprises en procédure de sauvegarde ? En effet, beaucoup de domaines viticoles, familiaux, affaiblis par la crise du secteur en 2019, du secteur en 2019, y ont eu recours. Dès lors, il devient important que le champ d'application du PGE soit étendu à ces entreprises, d'autant qu'une procédure de sauvegarde ne préjuge pas de la capacité de l'entreprise à rebondir, bien au contraire. Cette extension peut viser toutes les entreprises en sauvegarde, sans limite de date, puisque le droit des procédures collectives fixe expressément la durée maximale de la période d'observation, ce qui exclut, par essence, tout risque d'effet d'aubaine. Quel

Ces dernières sont considérées « à risque », car les crédits qui leur sont consentis par les banques ne peuvent être refinancés par la Banque centrale européenne, ce qui accroît la probabilité du refus du concours bancaire.

des personnes morales de droit étranger qui ont un intérêt stratégique pour notre pays ou pour des entreprises françaises.

Monsieur le rapporteur, je ne propose pas un dispositif ! Je demande un rapport sur ces questions, qui sont essentielles pour la défense de nos intérêts. Le monde d'après, ce ne sera pas une France derrière ses frontières et confinée

afin de favoriser durant la crise le renforcement en fonds propres des entreprises, et, d'autre part, de maintenir le bénéfice du dispositif de prêt garanti par l'État pour les seules entreprises procédant au versement de leurs dividendes

négatifs puissent prétendre au PGE. Avoir des fonds propres négatifs ne signifie pas que l'entreprise n'est pas saine et pérenne. C'est un indicateur qui est utilisé pour la solvabilité, mais qui n'est pas toujours le plus pertinent. Ce PLFR 2 est l'occasion de corriger cette inexactitude et de procéder à cette extension. Quel

et en accord avec la Fédération bancaire française, nous confirmerons, dans la foire aux questions qui pose notre doctrine, que les banques ne sont tenues à aucune vérification concernant ce critère de fonds propres. Elles peuvent donc prendre note du fait qu'il ne conditionne pas la validité de la garantie de l'État.

En outre, l'article 12 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 prévoit déjà la suspension des contrats de Cahors pour 2020, desserrant ainsi les contraintes sur la progression des dépenses de fonctionnement pour toutes les catégories de collectivités territoriales.

pour ne pas pénaliser les territoires et permettre aux collectivités territoriales de jouer pleinement leur rôle dans la reprise de l'activité économique dès la sortie de crise, il convient de proroger d'un an les délais d'engagement et de clôture des opérations d'investissement bénéficiant de subventions d'État.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

vise à renforcer l'article 12, dépourvu de tout caractère normatif et présentant des difficultés pratiques d'application. Dans sa rédaction actuelle, l'article 12 se limite à demander au Gouvernement la remise d'un rapport au Parlement dans les douze mois permettant d'évaluer le bon usage des ressources publiques par les entreprises soutenues. Il nous semble bien en deçà de l'ambition qu'il faut avoir en matière d'environnement et de climat. Nous comprenons qu'il faille faire vite au regard des conséquences économiques de la crise sanitaire.

des entreprises concernées. Si nous sommes favorables au renforcement de l'information du Parlement que nous proposera le rapporteur général dans quelques instants, nous demandons également un conditionnement de l'aide aux entreprises, nous demandons également un conditionnement de l'aide aux entreprises, afin que celles-ci s'alignent sur les objectifs de l'accord de Paris. Il serait incohérent, face à cette crise sanitaire et au regard du lien entre déclin de la biodiversité et émergence de maladies, de ne pas anticiper la crise écologique. C'est la raison pour laquelle nous suggérons de conditionner le sauvetage financier des entreprises à la simple publication, dans les douze mois, d'une stratégie interne de réduction de leur empreinte écologique et d'alignement sur l'accord de Paris. Il s'agit d'une mesure peu contraignante, mais qui remplit un double objectif : inciter les entreprises soutenues à se tourner vers l'avenir en se dotant d'une stratégie

que toute grande entreprise soutenue rende publique une évaluation de son empreinte carbone mesurant ses émissions directes et indirectes, une stratégie à même de réduire cette empreinte en en conformité avec les objectifs de l'accord de Paris, ainsi qu'un plan d'investissement et de transformation interne. Il s'agit de répondre aux légitimes inquiétudes

dispose : « L'Agence des participations de l'État veille à ce que ces entreprises intègrent pleinement et de manière exemplaire les objectifs de responsabilité sociale, sociétale et environnementale dans leur stratégie, notamment en matière de lutte contre le changement climatique.

et tout est fait pour que le Parlement ignore ce qu'en fera l'État. Voilà où en est la démocratie française

compte tenu de l'effort financier exceptionnel demandé aux Français, et à des fins de bonne utilisation des deniers publics, à rendre systématique le recouvrement des aides attribuées aux entreprises ayant des activités dans des paradis fiscaux.

français lorsqu'il s'est rendu compte qu'il avait des difficultés pour appréhender et accompagner la crise sanitaire ? Il a installé à côté du Président de la République un conseil scientifique,

pour faire face à la crise provoquée par l'épidémie de Covid-19. Le Gouvernement a mis en place une incompatibilité entre aide d'État et versement de dividendes pour le contrat de prêt garanti par l'État, qui prévoit une clause sur le sujet. pour les reports de charges et d'impôts. Dans la même logique, cet amendement tend à élargir ce dispositif aux entreprises concernées par le soutien prévu à l'article 4 du projet de loi, qui permet le sauvetage d'entreprises stratégiques.

En revanche, il est clair que nous avons systématiquement demandé à l'ensemble des entreprises de faire preuve d'une modération absolue sur le versement des dividendes et les rémunérations des dirigeants.

M. Emmanuel Capus. L'article 13 donne la possibilité au ministre de l'économie et des finances d'octroyer des avances remboursables et des prêts bonifiés aux PME stratégiques pour un territoire.

une subvention de fonctionnement global pour aider les associations à faire face aux adaptations rendues nécessaires par la crise sanitaire. Il est également possible, en dernier ressort, que l'autorité administrative

Je profite de la discussion de cet article, qui concerne l'assurance, pour rappeler que le groupe socialiste et républicain a déposé un amendement relatif à l'encadrement des frais bancaires en général. C'est devenu une question d'importance dans la crise que nous traversons.

être étudiée. La question des frais bancaires est essentielle, notamment pour toutes les familles et les personnes fragilisées durant cette période. Nous souhaitons que la majorité sénatoriale et le Gouvernement

et les agents économiques de leur territoire, qui font face à des situations difficiles avec la crise sanitaire liée au Covid-19. Leur implication sera particulièrement déterminante dans la mise en oeuvre des mesures arrêtées ou préconisées par le Gouvernement de protection sanitaire et le retour progressif à une activité « normale » de nos concitoyens. Cet amendement vise donc à imputer à la section investissement les dépenses des collectivités territoriales liées à la gestion de la crise du Covid-19.

au fonds national de solidarité. Afin de faciliter et d'amplifier les aides des collectivités locales, il conviendrait de ne pas limiter cette possibilité à ces seules contributions, mais de l'élargir à toutes les aides versées par les collectivités locales aux entreprises et aux associations qui exercent une activité économique dans le cadre de la crise sanitaire. Il importe notamment d'étendre cette possibilité aux fonds de solidarité territoriaux, qui sont en train d'être alimentés par les régions et par les EPCI. Cela leur permettrait alors de les

Mme la secrétaire d'État. Les crédits dédiés au fonds de solidarité pour les entreprises sont rehaussés de 2 milliards d'euros, compte tenu de l'amendement n° 207. 20 millions de crédits sont alloués à une prime exceptionnelle pour les assistants familiaux. Ces augmentations de crédits sont gagées par une réduction à due concurrence des crédits du programme « Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

L'impact sur le solde budgétaire de l'État est ainsi nul : le déficit est inchangé par rapport à la première partie s'établissant à 185,6 milliards d'euros.

Le scrutin est ouvert.